Entre 2012 et 2019, le nombre de bénéficiaires de l'AME de droit commun a déjà augmenté de 32 %, induisant une majoration des dépenses de près Ne

(AAH), L'AAH tend à se stabiliser en 2020, après deux années marquées par des revalorisations, qui doivent être saluées, même si elles se sont accompagnées- nous avions déjà eu l'occasion de l'expliquer

À cet égard, nous porterons un amendement visant à mettre en place un « minimum jeunesse ». Concernant le handicap et la dépendance,

Néanmoins, sont-ils suffisants au regard des enjeux ?

peut être saluée, le projet de loi de finances témoigne d'un réel soutien aux collectivités territoriales. Les crédits affectés à l'entretien et à la restauration des monuments n'appartenant pas